qui consentent des abandons de loyer à leurs entreprises locataires particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire. L'article 3 C prévoit notamment d'étendre la portée du dispositif voté par l'Assemblée nationale aux personnes morales de droit public telles que les établissements publics ou les collectivités territoriales et leurs groupements. En qualité de bailleurs, ces dernières pourront bénéficier d'un dispositif de compensation financière permettant de supporter le coût des abandons de loyers consentis.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, des dispositions ont été glissées dans cet article, et si nous n'avons pas eu le temps de déposer un amendement pour les contester, nous souhaitons tout de même interroger le Gouvernement et l'alerter au sujet de la modification de la perception de la taxe d'aménagement.

Le présent article introduit une modification de ces modalités de perception. En effet, les nouvelles dispositions proposées prévoient que cette taxe sera perçue par la commune à compter de la réception de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux.

décalent dans le temps le versement de la taxe d'aménagement- ce qui est bien regrettable -et, d'autre part, risquent de créer des contentieux que les services n'ont pas les moyens de gérer. Nous ne pouvons accepter une telle complexification de la perception de la taxe d'aménagement pour les communes.

dans un contexte de prix du foncier agricole comparativement plus faible en France que dans d'autres pays européens, sont responsables de l'artificialisation de 596 000 hectares de terres en dix ans.

qui n'atteignent pas un seuil minimal de densité de bâti. Le Gouvernement justifie sa suppression par le faible nombre de communes ayant souscrit au dispositif, et par conséquent, le faible rendement pour l'État de ce versement. Cette suppression n'est donc en rien motivée par une déficience du dispositif en tant que tel, mais bien par l'absence de volonté du Gouvernement de créer les conditions de sa réussite. C'est un dispositif facultatif proposé aux collectivités territoriales. De fait, très peu de communes ou d'EPCI le connaissent, car il n'a fait l'objet d'aucune promotion. l'État a supprimé le coefficient d'occupation des sols, rendant difficile la fixation d'un seuil minimal de densité par les collectivités. Plutôt que de créer des dispositifs fiscaux pour les supprimer quelques années après, l'État gagnerait en efficience s'il se donnait les moyens de leur succès. Le Gouvernement aurait ainsi tout intérêt à maintenir le versement pour sous-densité, à le promouvoir, voire à le rendre obligatoire, et surtout à apporter une aide administrative aux collectivités pour qu'elles puissent l'appliquer.

Le VSD répond à une volonté de maîtriser et de ralentir l'artificialisation des terres. C'est une conquête du Grenelle de l'environnement : sa

II-1277 visent à supprimer les dispositions tirant les conséquences de l'abrogation du versement pour sous-densité

Cet amendement vise à supprimer la demande d'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances toutes les mesures nécessaires à la refonte des taxes d'urbanisme faisant l'objet d'un transfert de gestion à la DGFiP.

ni du niveau d'imposition, ni des niveaux d'exonération, ni des règles d'affectation aux collectivités territoriales. L'article 44 a pour objet de permettre au Parlement de valider le schéma de transfert, afin de permettre à l'administration d'engager ces travaux complexes en toute sécurité. Un important travail a donc été réalisé pour inscrire dans la loi les principaux changements induits par la réforme et présenter ses objectifs et ses conséquences pour les redevables, mais aussi pour les collectivités territoriales. Le recours à une ordonnance pour organiser ce transfert, simplifier et requalifier les dispositions fiscales n'est pas inédit : le Parlement l'a validé pour les impositions sectorielles en loi de finances pour 2020. Un tel recours évite d'alourdir l'examen du projet de loi de finances de la discussion techniques. Le calendrier prévu permettra de consulter les collectivités territoriales, qui seront les premières bénéficiaires des gains de simplification et d'efficience permis par le transfert, de façon approfondie sur le texte. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut,

leur valeur n'est pas considérée comme étant à inclure dans l'assiette des cotisations sociales. En revanche, quand ces cartes sont utilisables à titre privé, elles constituent bien pour partie un avantage en nature.

prévoit que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux, l'Assemblée de Corse et le conseil régional de la peuvent exonérer de la taxe d'aménagement un certain nombre de secteurs d'activité comme les maisons de santé, les commerces de détail de moins de 400 mètres carrés ou les monuments historiques. La catégorie des hôtels, bars et restaurants ne figure pas dans ce périmètre d'exonérations. Or ces activités Or ces activités ont certainement été les plus durement touchées par la crise du covid, puisqu'elles ont été obligées de cesser pendant la durée des périodes de confinement et qu'elles auront connu six mois

des bars et de la restauration.

mesure d'exonération facultative n'aurait qu'un impact relativement marginal sur les établissements visés. Enfin, je tiens à rappeler que l'arsenal d'aides économiques a été amélioré et renforcé,

du Gouvernement ? La règle actuelle a pour conséquence de priver les usagers de l'utilisation de procédés électroniques de rédaction des actes. La mesure proposée par le sénateur Bargeton

Par ailleurs, les suppressions de postes qui sont envisagées entraîneront la fermeture d'un certain nombre de bureaux des douanes, qui assurent un rôle de contrôle, de recouvrement, mais également de conseil

en matière tant de conseil que de contrôle. Les entreprises savent que ce dernier volet est essentiel pour maintenir leur position compétitive dans un environnement économique tel que le marché unique européen.

À terme, la disparition du réseau des bureaux de proximité est programmée. Dans deux départements de la région Occitanie dont je suis élue- les Hautes-Pyrénées et la Lozère -, ces services publics ont été supprimés. Il s'agit souvent de petites structures, comptant entre trois et six agents, qui reçoivent et conseillent les opérateurs, mais effectuent également des contrôles de conformité, y compris dans les sociétés. Alors que la crise liée à la pandémie mondiale de covid-19 a mis en exergue l'impérieuse nécessité de retrouver, en France, une souveraineté industrielle, alimentaire et sanitaire, et tandis que l'urgence climatique devrait imposer une relocalisation généralisée de tout l'appareil productif, organiser l'inefficience du seul service qui est en mesure de procéder au contrôle physique des marchandises en mouvement non seulement est contre-productif, mais surtout porte gravement atteinte au seul principe censé sous-tendre l'action publique

Ensuite, des compensations sont prévues pour les effectifs de la douane qui seraient affectés par ce transfert. La douane connaît également un important processus de réorganisation, notamment pour faire face aux conséquences la DGFiP- elle l'a démontré avec le prélèvement à la source -est en mesure d'accueillir ce transfert. Chaque transfert s'accompagne d'une concertation importante entre l'administration et les acteurs économiques concernés pour faciliter la transition.

la DGFiP le recouvrement des recettes publiques et à transférer la gestion du droit annuel de francisation des navires (DAFN) à la direction des affaires maritimes, qui gère déjà la francisation.

par une société tête de groupe. Une telle définition conduit à exclure une grande partie du secteur du logement social. Par conséquent, en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le principe d'une dérogation au profit des acteurs du logement social que sont les sociétés de coordination et les organismes qui les détiennent,

à l'ensemble des sociétés comportant majoritairement des organismes HLM, des sociétés d'économie mixte (SEM) de construction et de gestion de logements sociaux et des SEM d'outre-mer. En effet, les entités des groupes d'organismes de logement social et les SEM d'outre-mer sont, en vertu de la loi,

surcoût de TVA de 20 % dans le cas où les actionnaires concernés mutualisent des moyens humains et matériels au sein de la filiale ou d'un groupement, alors que ce mouvement de regroupement et de mutualisation des moyens a été fortement encouragé, voire imposé, par la loi du 23 novembre 2018 portant

Le logement social fait partie de l'économie sociale et solidaire dans notre pays ; il importe de prêter une attention particulière à ce secteur, qui doit disposer des outils lui permettant de fonctionner dans les meilleures conditions.

le critère n'est pas adapté à certaines entités, eu égard à leur structure capitalistique ou à leur organisation particulière. Une série de présomptions a donc été prévue. De telles présomptions ne sont pas nécessaires quand les entités en cause sont susceptibles de satisfaire aux critères de droit commun pour caractériser un lien financier. Or la référence proposée au code de commerce, de l'amendement n° II-868 rectifié, implique une détention en capital ou en droits de vote. Elle s'appuie donc sur les mêmes critères que ceux actuellement prévus par le texte. La mesure proposée aurait pour effet d'introduire des critères de détention alternatifs dans un seul secteur économique. Cela peut nuire à la lisibilité du dispositif et rendre sa mise en oeuvre très complexe, notamment vis-à-vis de la Commission européenne, sans pour autant avoir la garantie de faciliter significativement la constitution d'un assujetti unique. Enfin, le Gouvernement est favorable à la mise en place d'une présomption de lien financier pour les sociétés de coordination, ce qui devrait permettre au secteur du logement social de bénéficier totalement du mécanisme de l'assujetti unique.

du code général des impôts (CGI) pour éviter la double imposition. Cette proposition paraît tout à fait compatible avec la directive TVA- l'amendement devrait donc passer ! -, qui réserve le régime des groupements autonomes de personnes aux activités d'intérêt général listées dans son article 132.

à l'aide et à la sécurité sociale. La

cas où, cet amendement de repli visant à permettre au secteur du logement social de continuer à utiliser le régime de l'article 261 B du code général des impôts jusqu'au 31 décembre 2024.

nécessite un examen au cas par cas. Or votre amendement pose un principe général d'exonération. La mise en place du régime du « groupe TVA » au sein de cet article 45 est de nature à limiter les impacts de la suppression du dispositif des groupements autonomes de personnes (GAP) en neutralisant la facturation de la TVA pour les opérations effectuées entre les membres et à apporter de la sécurité juridique

avec un taux élevé de pauvreté des ménages, autour de 20 %., 80 % des ménages sont susceptibles d'être éligibles à un logement social. Il est, par conséquent, difficile de faire face à cette forte demande. En outre, la pression immobilière et foncière sur l'île incite davantage à la construction de résidences luxueuses que de logements sociaux. Depuis les années 2000, la Corse, compte tenu de son insularité qui entraîne, notamment, un surcoût des matériaux de construction, bénéficiait, comme les outre-mer, d'un différentiel de taux de TVA pour la construction de logements sociaux par rapport au continent. des différentes variations de taux selon les années en France métropolitaine, la Corse a toujours bénéficié d'un taux réduit à 5,5 %. Néanmoins, depuis le 1 janvier 2018, le taux réduit de TVA a été relevé à 10 % partout en France, hors outre-mer. Ainsi, contrairement aux autres territoires insulaires, la spécificité n'est donc plus prise en compte en Corse. Ce relèvement brutal du taux de TVA s'avère particulièrement lourd à gérer pour les bailleurs sociaux, notamment pour l'office public de l'habitat de la collectivité de Corse (OPH). Cela représente, pour ce dernier, 1 million d'euros de surcoût à puiser sur les fonds propres pour les seules opérations en cours, soit 173 logements en construction. De plus, la vulnérabilité à la baisse des apparaît également plus marquée pour la Corse : tous les locataires de l'OPH de Corse sont éligibles à l'APL. Il faut ajouter à cela la baisse drastique des aides à la pierre ou encore la perte pour la Corse du taux préférentiel sur le règlement national de l'Agence (ANRU). Notons également l'impossibilité de fusionner les organismes publics en Corse- il s'agit d'une exception à la loi ÉLAN -, que la majorité territoriale corse ne demandait pourtant pas et qui aurait permis d'effectuer des économies d'échelle.

rappeler. La construction de logements sociaux bénéficie déjà d'un taux à 5,5 % depuis la loi de finances pour 2019 concernant les constructions neuves financées par le prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) ou par le prêt locatif à usage social ainsi que dans les quartiers faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville.

L'amendement proposé remet en cause l'orientation du Gouvernement consistant à cibler spécifiquement les logements des personnes aux revenus les plus modestes, les logements PLAI,

Il s'agit de faire bénéficier les CD, les vinyles et les téléchargements légaux d'un taux de TVA à 5,5 % à compter du 1 janvier 2022, près de dix ans après l'application d'un taux réduit de TVA pour les livres audio. L'activité des labels reste encore très dépendante des achats physiques, qui représentent 37 % des ventes de musiques enregistrées. Le confinement lié au covid a durement atteint le secteur

Le risque d'effet d'aubaine pour les productions étrangères est d'ailleurs particulièrement faible, puisque 19 des 20 meilleures ventes sont des productions locales chantées en français.

néanmoins, il y a une difficulté de comptabilité avec le droit communautaire. C'est la raison pour laquelle j'émets, comme en première partie, un avis défavorable.

dans la doctrine fiscale ou par rescrit est envisageable, voire intéressante, pour clarifier les règles applicables aux cartes. Par

d'adoption, qui sera publiée avant la fin de l'année. Par ailleurs, ces vaccins devront répondre aux exigences prévues par le droit européen et le droit national. Un taux de TVA à 0 %, appliqué de manière provisoire à ces vaccins essentiels à notre stratégie de lutte contre la pandémie de covid-19,

La condition de grade actuellement prévue est une surtransposition du droit de l'Union européenne. La La mesure proposée par le sénateur Iacovelli et défendue par le sénateur Bargeton permettra de renforcer la lutte contre la fraude en matière de tabac et de préserver les intérêts du Trésor. L'avis est donc favorable.

a démontré que les paramètres actuels du dispositif ne permettaient pas réellement à la dépense publique d'être totalement efficiente ni de participer vraiment efficacement à la lutte contre l'artificialisation des sols. Pour résumer, le Gouvernement s'est engagé à proroger

l'après-2023, mais je préfère le marbre de la loi. Vous nous avez trop habitués au « en même temps », à ce double discours qui consiste à nous dire : « Vous avez raison, mais on verra plus tard. » Puisque nous avons raison, nous allons voir tout de suite !

les primo-accédants ruraux- ce sont souvent des ménages de jeunes -sont pénalisés au titre de la quotité. En effet, en zones A et B1, pour un couple de jeunes qui veut construire, le prêt à taux zéro peut couvrir 40 % du coût de la construction,

qui crée une inégalité territoriale et une rupture d'égalité de traitement entre les Français. C'est justement dans les zones moins tendues, où les prix d'acquisition sont encore accessibles aux ménages, que le PTZ prend tout son sens. C'est la raison pour laquelle notre amendement a pour objet de supprimer le facteur de localisation du logement dans la définition de la quotité du coût total de l'opération.

On évoque très régulièrement ceux qui ne peuvent accéder au logement. Si l'incitation à l'accession à la propriété est plus soutenue, cela aidera à libérer des logements locatifs publics et à résoudre ce problème sociétal

à l'accession sociale à la propriété, d'un montant de 15 000 euros, versée par les établissements de crédit et les sociétés de financement, un mécanisme de crédit d'impôt. Bien évidemment,

depuis 2001, la part des dépenses de logement dans les revenus est passée de 31 % à 42 % pour les 10 % les plus pauvres, tandis qu'elle a évolué de 9,8 % à 10,8 % pour les 10 % les plus riches. Rapporté aux revenus, le logement coûte donc quatre fois plus cher pour les pauvres, et son poids est en constante augmentation depuis 1980. Compte tenu des prix de l'immobilier, le quart des habitants les plus pauvres qui souhaitent accéder à la propriété doivent consacrer, en moyenne, près de la moitié de leur budget au logement, et les plus modestes deviennent de moins en moins souvent propriétaires. Entre 25 et 44 ans, près d'un ménage sur deux est propriétaire, mais la

supplémentaires. En outre, pourquoi faire intervenir les banques dans ce qui est en fait une aide de l'État pour les accédants à la propriété ? Les choses sont différentes pour le prêt à taux zéro : les banques sont dans leur rôle, puisque ce sont elles qui accordent un prêt.

Premièrement, il vise à prolonger de trois ans le dispositif expérimental habilitant les sociétés de tiers-financement à distribuer l'écoprêt à taux zéro.

Dans un contexte de recherche d'amélioration de la performance énergétique des logements, les sociétés de tiers-financement sont des outils innovants encouragés tant par la loi ALUR que par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Les projections issues du rapport du plan urbanisme construction architecture (PUCA) font apparaître des gains énergétiques multipliés par cinq entre 2020 et 2026 s'agissant des chantiers suivis par les sociétés de tiers-financement. Pour mesurer à plein les effets de cette expérimentation, cet amendement vise à prolonger sa durée de trois années supplémentaires et à étendre son champ géographique à l'ensemble du territoire.

ne visent qu'à prolonger l'expérimentation jusqu'en 2024. Je rappelle que cette expérimentation a pour objet de tenter de « sauver », en quelque sorte, ce dispositif, victime d'une forme de complexité administrative et d'un manque d'attractivité pour les banques, dont, il faut le reconnaître, la rénovation énergétique est loin d'être le métier. Les établissements de tiers-financement, qui, eux, sont beaucoup plus spécialisés dans ce type de travaux que les banques, pourraient, de mon point de vue, faciliter la distribution de ce produit. Toutefois, à ce stade, une généralisation me paraît prématurée. Il convient d'attendre le résultat de l'expérimentation, sur laquelle le Gouvernement doit remettre un rapport d'évaluation au plus tard le 30 septembre de l'année prochaine.

résolution (ACPR) pour distribuer les prêts sont soumises à un régime de supervision trop peu exigeant pour que nous ne doutions pas de l'opportunité de les autoriser à distribuer les écoprêts à taux zéro. De fait, nous ferions peser un risque financier sur les collectivités territoriales. Le Gouvernement pense aussi qu'il est préférable d'attendre les conclusions de l'expérimentation en cours

grandes consommatrices d'énergie, c'est-à-dire « dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée

d'un système de management de l'énergie et à l'adhésion de l'exploitant à un programme de mutualisation de bonnes pratiques, à compter du 1 janvier 2022. La commission propose d'aller

en soumettant le bénéfice de l'avantage fiscal à la condition de valorisation de la chaleur fatale par l'exploitant du centre de stockage de données numériques.

analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid

Cette exonération étant facultative, la perte de recettes qui en résulte relève de la libre administration des collectivités concernées. En outre, cette exonération peut permettre de garantir l'équilibre du service public de la chaleur, sans faire supporter aux usagers le poids des impôts locaux dans le tarif sa répercussion sur la facture du consommateur. Le développement attendu des réseaux de chaleur dans les années à venir est à souligner : la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif, à l'horizon 2030, de multiplication par cinq de la quantité de chaleur renouvelable et de récupération par rapport à 2012. La trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l'énergie confirme cette volonté.

2023. Dans ce contexte, il est nécessaire de soutenir fiscalement les réseaux de chaleur utilisant de la chaleur renouvelable et de récupération pour atteindre les objectifs fixés.

La taxe foncière sur les propriétés bâties est un impôt dû à raison de la détention d'un bien immobilier, quelle que soit l'utilisation qui en est faite. Par conséquent, les exceptions à ce principe doivent être limitées et justifiées. Par ailleurs, le Gouvernement a fait le choix de privilégier des outils plus ciblés comme le fonds chaleur, qui soutient notamment les réseaux de chaleur liés aux projets de production d'énergie renouvelable pour permettre à ces technologies d'être économiquement compétitives par rapport aux installations utilisant une énergie conventionnelle. La grande

amendement vise à prolonger cet avantage fiscal pour les chefs de très petites entreprises, selon les critères européens de la définition de la microentreprise, qu'ils soient assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

d'un sujet important auquel le Gouvernement est particulièrement sensible. Les entreprises bénéficient déjà d'un certain nombre de dispositifs d'aide à l'acquisition et à l'installation de systèmes de recharge pour véhicules électriques- à la prime Advenir, qui couvre les coûts de fourniture d'installation, à hauteur de 40 % en 2020 et 30 % en 2021, des points de recharge sur parking privé à destination des flottes

000 bornes dès 2021, contre 2022 initialement. La loi prévoit aussi une obligation d'équipement de systèmes de recharge pour les bâtiments neufs ou les bâtiments rénovés à usage principal industriel ou tertiaire qui comportent un parc de stationnement

Gremillet, cosigné par de nombreux sénateurs, tend à compléter le rapport annuel sur l'impact environnemental du budget d'une évaluation de l'incidence du plan de relance sur l'atteinte de nos objectifs énergétiques et climatiques. En effet, un an après l'adoption de la loi Énergie-climat, l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, adopté dans un esprit de consensus par l'Assemblée nationale et le Sénat, ne doit pas être un vain mot. Tout au contraire, le Gouvernement doit allouer des moyens budgétaires et fiscaux en regard des objectifs énergétiques et climatiques fixés par le législateur et veiller à leur mise en oeuvre concrète auprès des acteurs économiques et des collectivités territoriales. Il est donc nécessaire de compléter l'information du Parlement pour s'assurer que les 30 milliards d'euros du plan de relance alloués à l'écologie, et singulièrement les 15 milliards d'euros

vise à compléter le rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État, avec une évaluation de l'incidence du plan de relance sur l'atteinte de nos objectifs énergétiques et climatiques, en particulier sur la stratégie nationale bas carbone. Ce rapport présente, outre la cotation des dépenses de l'État et du plan de relance, selon la méthode du « budget vert », une évaluation des moyens financiers publics et privés en faveur de la transition écologique et du climat. Ce rapport a vocation à se pérenniser, et il n'apparaît pas véritablement opportun de prévoir un développement dédié au plan de relance,

Cet amendement de notre collègue Gérard Longuet vise à favoriser les investissements réalisés par les entreprises ayant pour objet la réduction de leur consommation d'énergie et financés par le biais des certificats d'économies d'énergie, Actuellement, sur le plan comptable, les CEE perçus par les entreprises sont, sur option, soit immédiatement comptabilisés en produit, soit inscrits au passif du bilan en subvention d'investissement et rapportés au résultat tout au long de la période d'amortissement des installations réalisées. L'option d'étalement permet à la société de rapporter tout au long de la durée d'utilisation de l'installation à la fois la quote-part annuelle de produit de CEE et la quote-part annuelle d'amortissement de l'installation financée par ces CEE. Sur le plan fiscal, la faculté d'étalement de la fiscalisation des subventions est limitée par l'article 42 du du code général des impôts aux subventions accordées uniquement par « l'Union européenne, l'État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public ». Or les CEE sont attribués par des organismes privés dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale. Ils ne sont donc pas éligibles à cet étalement. actuelle, les CEE sont imposés immédiatement sur l'exercice comptable au cours duquel ils sont acquis. Il en résulte un surcoût immédiat qui ne favorise pas la trésorerie des entreprises qui investissent dans la réduction de leur consommation énergétique. Il est contre-productif d'aider les entreprises à financer ces installations économes en énergie, tout en reprenant immédiatement par l'impôt 28 % de cette aide dès son attribution. Afin de favoriser ces investissements, il est proposé une concordance des règles comptables et fiscales en matière de CEE pour permettre un lissage de l'imposition de ces subventions. CEE pourraient alors, sur option, ne pas être imposés sur le seul exercice de leur attribution, mais être imposés de manière échelonnée comme les subventions publiques. Il est proposé, à compter des exercices clos le 31 décembre 2020, de compléter le premier alinéa du 1 de l'article 42 du code général des impôts en insérant, après les mots «

une extension significative du dispositif d'imposition prévu en matière de subventions publiques. L'extension de ce dispositif à des financements attribués dans le cadre des

des demandes similaires. Les certificats d'économies d'énergie reposent sur une obligation triennale de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d'énergie, dits les « obligés derniers sont ainsi incités à promouvoir activement l'efficacité énergétique auprès des consommateurs d'énergie. Les CEE sont attribués par les services du ministère chargé de l'énergie, sous certaines conditions, aux acteurs éligibles, « obligés » par d'autres personnes morales non obligées réalisant des opérations d'économie d'énergie. Ces certificats sont également acquis auprès d'acteurs privés ayant mené des actions d'économies d'énergie. L'économie générale de ce dispositif repose donc sur des transactions entre acteurs privés ; c'est d'ailleurs tout son intérêt. Le dispositif d'étalement des subventions publiques d'équipement constitue une dérogation au principe selon lequel un produit est imposable au titre de l'exercice au cours duquel il est acquis. est acquis. Il se justifie pour autant que le financement constitue une aide publique à l'investissement. Il n'a donc pas vocation à s'appliquer aux versements réalisés dans le cadre des certificats d'économies d'énergie, qui n'ont pas nécessairement la nature de subventions d'équipement et donnent lieu à des transactions entre personnes privées.

sur le sujet, notamment celui du Conseil des prélèvements obligatoires, qui, à ce jour, fournit une vision complète de la fiscalité environnementale française.

contre 28 000 euros pour un soutien aux investisseurs institutionnels, soit 35 % de moins dans ce dernier cas, pour une qualité généralement supérieure. Cinquièmement, une incitation insuffisante en termes de qualité des logements construits et de qualité de la gestion des copropriétés en résultant.

La ministre chargée du logement a indiqué, lors de la présentation de la mission « Cohésion des territoires », que le Gouvernement prévoyait de présenter une réforme

d'envisager des dispositifs alternatifs plus efficients et plus économes, impliquant notamment une intervention accrue des « zinzins Toutes ces évolutions témoignent de la détermination claire et totale du Gouvernement à améliorer l'emploi des moyens alloués à la politique publique en faveur du logement, comme l'a d'ailleurs rappelé Emmanuelle Wargon,

Supprimer le Pinel d'un trait de plume, c'est la garantie absolue que le marché de l'immobilier, qui n'est pas en grande forme, c'est le moins que l'on puisse dire, s'effondre. On ne peut donc pas faire cela.

en échange d'une réduction fiscale. Les particuliers viennent donc en aide à l'État pour répondre au problème du logement et favoriser des travaux.

qui limite, à compter du 1 janvier 2021, le bénéfice du Pinel aux bâtiments d'habitation collectifs. En supprimant cet article, vous ne supprimeriez pas ce qui a été voté en projet de loi de finances pour 2020.

L'article 164 de la loi de finances pour 2020 a en effet introduit la possibilité d'étendre le bénéfice de cette réduction d'impôt à la vente de logements neufs dans certaines communes ou parties de communes bretonnes situées en zones B2 et C. La fin de cette expérimentation est prévue pour le 31 décembre 2021. Or celle-ci n'a pu être lancée que tardivement, puisque l'arrêté préfectoral redessinant la cartographie de l'éligibilité à la réduction d'impôt n'est applicable que depuis le 31 mars 2020. Ce retard, amplifié par les conséquences de la crise sanitaire, affectera sans nul doute le bilan de l'expérimentation, le rapport de l'État sur le sujet devant être remis au Parlement avant le 30 septembre 2021. Dans le même temps, les collectivités délégataires des aides à la pierre ont travaillé activement avec la région Bretagne et les services de l'État afin de répondre aux besoins en logements intermédiaires locatifs, en forte croissance sur le territoire. Le monde économique a également participé à l'ensemble de cette démarche et soutenu les mesures mises en place sur un territoire breton reconnu de longue date pour sa capacité à tenir ses engagements. C'est d'ailleurs tout l'intérêt et toute la richesse de l'expérimentation que d'intégrer des spécificités territoriales en s'appuyant sur les dynamiques locales dans le respect des grandes orientations nationales. Dans un contexte de relance de la construction et de pression locative accrue, nous proposons donc, par cet amendement, d'aligner le terme de cette expérimentation sur celui du dispositif national, donc de le porter au 31 décembre 2022.

Estrosi Sassone. L'acquéreur d'un logement neuf ne peut bénéficier de la réduction d'impôt Pinel que si ce logement est achevé dans un délai de trente mois à compter de la signature de l'acte authentique d'acquisition. Ce délai permet théoriquement de protéger les acquéreurs et de maintenir le maître d'ouvrage sous tension afin qu'il respecte l'échéance légale. Il présente toutefois deux défauts : il méconnaît, d'une part, la réalité des programmes immobiliers, qui nécessitent très souvent, par leur complexité, plus de trente mois ; d'autre part, il ne ménage aucune souplesse : la seule option offerte par la pratique administrative consiste à demander une prorogation aux services fiscaux, qui n'en accordent que de façon discrétionnaire et dans des cas très limités : force majeure ou recours contentieux. Il paraît donc souhaitable d'assortir ce délai de trente mois d'une forme de souplesse en ouvrant aux contribuables la faculté de demander aux services fiscaux le bénéfice d'une prolongation de délai pour une période d'un an renouvelable. Cette procédure, encadrée par le pouvoir réglementaire, est bien connue des opérateurs comme de la DGFiP, Cette modification aurait pour effet de simplifier le mécanisme des trente mois, d'améliorer la sécurité juridique et de protéger les consommateurs.

Cette restriction s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 1 janvier 2021. Cet article soulève une double difficulté. Une difficulté de définition, tout d'abord : à un mois de l'échéance, l'incertitude demeure sur ce que recouvre précisément la notion de logement collectif. Une difficulté de calendrier, ensuite : des projets de construction de logements collectifs lancés avant le vote de la loi de finances pour 2020 ont vu leur commercialisation gravement perturbée par l'épidémie de covid-19, de sorte qu'une partie de ces biens risque de ne pas pouvoir être vendue à des investisseurs Pinel avant le 31 décembre, sans pour autant pouvoir trouver d'acquéreurs-accédants à la propriété. L'objet du présent amendement est donc de reporter de six mois l'application de la restriction issue de la loi de finances pour 2020. Ce report permettrait aux services fiscaux, d'une part, de préciser la portée de la mesure par la définition des « bâtiments d'habitation collectifs ». Serait ainsi reconstitué un délai suffisant entre la clarification de la mesure et son entrée en vigueur, le délai d'un an initialement prévu par le législateur ayant été de fait neutralisé par l'absence de définition certaine. La publication de l'instruction fiscale, en dissipant l'imprécision qui entoure la notion de « bâtiments d'habitation collectifs », protégerait les investisseurs particuliers du risque fiscal né de l'incertitude dans laquelle ils sont aujourd'hui

Par ailleurs, la doctrine fiscale admet déjà des prorogations du délai en cas de force majeure, par exemple lorsqu'un arrêté municipal empêche la poursuite d'un chantier de construction ; il existe un rescrit fiscal en ce sens.

je rappelle deux choses : premièrement, le PLF 2015 avait modifié la date de début du délai en substituant à la date de début de chantier la date de fin de chantier ou de mise en commercialisation ; deuxièmement, l'ordonnance que nous avons prise au mois de mai neutralise la période d'état d'urgence sanitaire du printemps dans le calcul du délai, ce qui nous paraît répondre au moins en partie à l'attente ici formulée. L'avis est donc défavorable. Je mets

l'avis du Gouvernement ? Il s'agit d'une mesure qui a été intégrée dans le texte sur l'initiative du Gouvernement, avec un certain nombre d'aménagements, notamment le poids retenu et le fait d'exclure

est l'intérêt de notre industrie automobile ? C'est la question soulevée au travers de cette série d'amendements et de cet article 45. Si les mots « développement durable » ont un sens, s'ils sont autre chose qu'une formule de communication, il me semble que l'intérêt durable de nos constructeurs n'est pas de prolonger encore un peu plus cette dérive à courte vue qui consiste à produire du SUV, toujours plus de SUV, et à déployer tous les artifices publicitaires pour entretenir cette frénésie de consommation de grosses voitures.

C'est d'ailleurs dans le même état d'esprit que j'ai proposé au Sénat d'augmenter de 500 millions d'euros les crédits de la prime à la conversion dans le cadre du plan de relance. La création d'un prêt à taux zéro d'un prêt à taux zéro spécifique pour l'achat d'un véhicule propre va dans le bon sens. C'est une mesure particulièrement bienvenue.

Compte tenu de cette situation et de l'importance qu'il y a à donner à la CNCTR toute la crédibilité qu'elle mérite sur le contrôle de l'intimité

en donnant à la CNCTR la possibilité et le mandat non pas de remettre un avis au Premier ministre, comme elle le fait pour les questions de renseignement, mais une autorisation d'accéder aux données de connexion. Quel

et d'impartialité : le contrôleur sera un membre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation nommé pour quatre ans non renouvelable, et il ne pourra être mis fin à ses fonctions. Il s'agit d'un dispositif déjà éprouvé, qui existe pour l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de la concurrence.

procédure que vous proposez est d'une certaine manière disproportionnée. Elle serait lourde, coûteuse et pourrait engorger la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

On ne peut pas non plus dans un projet de loi de finances traiter d'un sujet qui ne relève pas du dispositif de l'article 34 de la LOLF, mais qui est beaucoup plus large, puisqu'il s'agit des libertés et du contrôle de l'accès aux données de connexion de l'ensemble des Français. Nous avons créé pour cela la CNCTR.

Elles organisent le traitement fiscal et comptable des opérations de prêts de titres. Elles reprennent à l'identique les dispositions du code monétaire et financier, qui prévoient le traitement comptable de ces opérations, dans le but d'assurer leur neutralité fiscale et de garantir que le traitement fiscal suive le traitement comptable préconisé.

de disposer de l'évaluation que nous avons prévue, notamment sur le périmètre des aviseurs. Mon propos n'est pas de remettre en cause le système des aviseurs, au contraire, puisqu'il a démontré son efficacité. Il faudra même certainement le renforcer et mieux l'encadrer. Allons néanmoins au bout de l'expérimentation avant de décider quoi

La première version du PLF à l'Assemblée nationale prévoyait, aux termes d'une proposition de Mme Peyrol notamment, la création d'un observatoire en charge de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale.

j'ai eu l'occasion de réunir, il y a quelques semaines, les attachés douaniers dont la France dispose dans différentes ambassades, notamment au sein de l'Union européenne, pour appeler leur attention sur ces questions d'échanges, de conventions et

Sur le premier point, il me semble que, pour toute créance, les douanes disposent bien d'un délai précis pour agir. Pour interrompre la prescription, le procès-verbal doit intervenir dans le délai prévu de trois ans à dix ans selon les cas. Sur le second point du dispositif de l'amendement, même si le procès-verbal interrompt la prescription dans le cadre du droit de reprise sur les ressources de l'Union européenne, il est bien précisé que ce droit de reprise n'est interrompu que dans une limite de dix ans, ce qui est conforme au droit de l'Union. Le Gouvernement pourrait-il nous apporter des précisions sur ces deux points, ainsi que sur la conformité au code des douanes de l'Union de l'interruption du délai de prescription par un procès-verbal ? Quel est l'avis du Gouvernement ? Le droit de l'Union européenne- je fais référence à l'article 103 du règlement 952/2013 du Parlement et du Conseil du 9 octobre 2013 -prévoit un délai de reprise de trois ans. Il permet aux États membres de le porter entre cinq et dix ans, conformément aux dispositions du droit interne de chaque État, lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives. Dès lors que les infractions douanières ont un caractère pénal, l'article 354 du code des douanes prévoit un délai de reprise de cinq ans, qui ne peut être interrompu au-delà de la dixième année qui suit celle au cours de laquelle les droits sont dus. Cette disposition, qui aménage la possibilité d'un délai de reprise de dix ans maximum, est donc conforme au droit de l'Union. Par ailleurs, la possibilité d'un délai de reprise de dix ans aménagé par le code des douanes, dès lors que cette interruption ne permet pas de dépasser le délai de dix ans, nous paraît être clarifiée par le I de l'article 46 du projet de loi de finances pour 2021. Enfin, Enfin, j'ajoute que la possibilité d'interrompre le délai de reprise par la notification d'un procès-verbal doit être maintenue. Elle est conforme au droit de l'Union et permet surtout de sécuriser

nous avions relevé à 1 000 euros le plafond pour lequel il est possible de faire un don à des associations d'aide aux personnes en difficulté, en bénéficiant de 75 % de réduction d'impôt.

un déplafonnement jusqu'à 1 000 euros pour l'année 2020. Nous faisons tous le constat que la crise est en train de s'approfondir et les grandes associations, comme le Secours populaire et le Secours catholique, nous ont alertés au sujet de la multiplication de la pauvreté.

et des échanges entre le Premier ministre et les associations du secteur, le Gouvernement est ouvert, et même favorable à la prorogation de ce dispositif pour l'année 2021. Encore

il faut reconnaître que l'inquiétude peut créer une baisse de la générosité. Cette mesure est donc un signe important à donner dans cette période de très grave crise sociale. Je veux aussi dire qu'une politique contre la pauvreté ne peut pas se résumer à cet amendement, aussi utile soit-il. J'entends les propos du Premier ministre, notamment lorsqu'il affirme vouloir lutter contre la pauvreté. Il serait temps de passer à des actes beaucoup plus massifs

Il a pour objet de prévoir l'autorisation préalable de l'administration fiscale pour les déductions qui concernent des dons ou des legs à des organisations

Je rappelle qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts, les dons consentis aux associations cultuelles ouvrent droit à la réduction d'impôt, qu'il s'agisse de legs prévus au testament du donateur, de donations du vivant du donateur ou de dons manuels.

domiciliées à l'étranger et qui déclarent sur l'honneur qu'il leur est impossible d'ouvrir un compte de dépôt dans l'espace unique de paiement en euros.

est à Mme Isabelle Briquet. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à mettre en place un dispositif du type « budget participatif » à l'échelon du pays à partir d'une fraction des recettes de l'impôt sur le revenu. Concrètement, les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu auront la possibilité d'affecter 5 % de leur impôt à une mission budgétaire. Ce choix devra s'opérer au moment de la déclaration de revenus. Concrètement, le contribuable devra cocher la case de loi de finances de l'automne suivant devra tenir compte de la ventilation de la fraction d'impôt sur le revenu par mission, afin de s'assurer que les choix des contribuables sont respectés.

à 74,936 milliards d'euros. Ce montant, qui correspondrait à 1,4 % des recettes fiscales nettes de l'État en 2021, ne mettrait donc pas en péril l'équilibre global du budget ni la répartition des crédits par mission. Il est évident que le dispositif de cet amendement est perfectible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas vocation à s'appliquer avant 2024. Ce délai permettra au Gouvernement de remettre un rapport sur le fondement duquel le dispositif pourrait être revu. Cet amendement a un objet clair et à la pertinence incontestable : renforcer le consentement à l'impôt, qui a fortement reculé ces dernières années. prenons modèle sur les budgets participatifs mis en place par certaines collectivités, comme les villes de Rennes et de Paris, ou le département des Landes. Nous pensons qu'il permet d'éviter un écueil : l'opposition entre démocratie représentative

l'équilibre, mais également l'universalité. Le principe d'universalité implique que l'ensemble des recettes assure l'exécution de l'ensemble des dépenses. L'adoption

Le prélèvement à la source est une réforme ambitieuse, qui a été engagée durant le précédent quinquennat pour garantir davantage de justice fiscale et de fluidité dans le recollement de l'impôt, et de lisibilité pour nos concitoyens.

la problématique d'une imposition basée sur le foyer fiscal, et non sur l'individu. Cette question se pose dans un contexte où la France demeure l'un des rares pays développés à appliquer une telle logique d'imposition. un rapport, qui traiterait de la possibilité d'élargir le dispositif du prélèvement à d'autres impositions. La question de la mise en place d'un système global fondé sur le prélèvement à la source, et incluant la possibilité de mettre en oeuvre

Je suis défavorable à cet amendement, qui vise à remettre en cause la place du foyer fiscal dans le système français, afin de

Monsieur Blanc,

parole est à Mme Laurence Cohen. Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi est chargé de l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi et répond aux besoins de recrutement des entreprises. L'article 46 autorise l'accès au fichier des contrats de capitalisation ou des placements de même nature aux agents de Pôle emploi, afin de leur permettre de mieux détecter les situations frauduleuses. Les informations transmises par les entreprises le sont à la direction générale des finances publiques d'assurance vie (Ficovie). Selon le type de contrat ou de placement, l'administration fiscale indiquera notamment la nature et la date du contrat ou du placement, les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile des assurés. Aujourd'hui, seuls les agents les agents habilités des finances publiques et des organismes de protection sociale, ainsi que les notaires peuvent consulter ce fichier. Les agents de Pôle emploi peuvent déjà avoir accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés et au fichier des données de l'immobilier. amendement du Gouvernement, reprend une proposition de la Cour des comptes pour améliorer la lutte contre la fraude. Je veux faire remarquer la différence de traitement entre le contrôle des prestations sociales et l'absence même de contrepartie pour les entreprises. Sur le fond, cet article pose une véritable question en autorisant les agents de Pôle emploi à accéder aux fichiers des contrats de 38 millions de personnes.

enfin, en autorisant les agents de Pôle emploi à accéder à ces fichiers, il me semble que l'on dépossède la direction générale des finances publiques d'une mission pour laquelle elle dispose d'agents formés.

Il vise à accorder aux indépendants le même abattement forfaitaire de 10 % qu'aux salariés, moyennant l'exclusion du calcul du résultat catégoriel imposable des dépenses couvertes par l'abattement forfaitaire ou la déduction des frais réels. Le contribuable déclarant lui-même son revenu, contrairement aux salariés dont les revenus sont déclarés par les employeurs, il est indispensable de conditionner le bénéfice de ce dispositif à l'adhésion à un organisme de gestion agréé- on a déjà eu ce débat précédemment aux services d'un professionnel de la comptabilité, afin de s'assurer que les dépenses ne sont pas déduites deux fois. La perte de recettes pour le budget de l'État devrait être en partie compensée par les recettes issues des cotisations sociales.

Je suis défavorable à ces amendements, qui mélangent en réalité deux débats distincts sans d'ailleurs, me semble-t-il, répondre aux difficultés réelles soulevées. En effet, leurs auteurs proposent d'étendre aux travailleurs indépendants la déduction des frais professionnels dont bénéficient les salariés. Or, pour les indépendants, l'imposition du revenu correspond à leur activité professionnelle, ce qui permet de tenir compte des charges exposées dans ce cadre. Par ailleurs, vous proposez également de conditionner cette mesure à l'adhésion à un organisme de gestion agréé, par mesure de repli par rapport à la suppression de la majoration prévue à l'article 7 du projet de loi de finances.

ne relève pas de la loi de finances toute disposition ne concernant ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties, ni encore la comptabilité de l'État. Or les dispositions du présent article ne paraissent relever d'aucune de ces catégories.

Cette fermeture a été et reste un traumatisme pour les habitants de la zone et les 830 salariés licenciés dans le mépris le plus total par l'actionnaire Glencore.

à traiter sur place ; 45 kilomètres carrés de terrain durablement pollués au plomb tout autour. En 2015, la préfecture du Pas-de-Calais a classé une partie de ce territoire en périmètre d'intérêt général, essentiellement sur les communes de Courcelles-lès-Lens, Évin-Malmaison et Noyelles-Godault, avec un encadrement strict des autorisations concernant les travaux et l'occupation des sols, faute de pouvoir mener une véritable dépollution.

qui s'y était pourtant engagé. Or, vous le savez, mes chers collègues, cette année 2020 n'a pas été la plus simple pour nos concitoyennes et nos concitoyens : une partie d'entre eux n'a pas relevé la subtilité administrative qui leur impose de déclarer annuellement auprès du trésor public qu'ils vivent toujours sur une terre polluée pour des décennies. Les contribuables en question ont donc vu leur impôt foncier doubler cette année par rapport à l'année précédente, suscitant un vent de panique et une incompréhension. Notre amendement a pour seul objet de simplifier cette démarche en la rendant automatique pour les propriétaires qui restent sur place, tant que les sols resteront pollués. Quel

Si l'obligation de déclaration annuelle semble effectivement excessive à mes yeux, je solliciterai tout de même l'avis du Gouvernement

est une victoire de l'optimisme sur l'expérience, monsieur le ministre. Il a pour objet de généraliser la procédure de flagrance fiscale qui est, pour le moment, limitée.

Je rappelle que la procédure de flagrance fiscale permet aux agents des finances publiques de dresser un procès-verbal des faits frauduleux qu'ils ont été amenés à constater. Ce procès-verbal permet notamment la prise immédiate de mesures conservatoires sans autorisation préalable du juge. Il est donc logique de circonscrire strictement son champ d'application. La commission est défavorable

Si l'on pousse plus loin l'analyse, on se rend compte que cette trésorerie a été artificiellement consolidée en un seul ensemble, alors qu'elle est divisée en plusieurs fonds, dans le respect des obligations réglementaires, et qu'elle était déjà largement engagée.

article 47, vous prenez de l'argent destiné à la construction pour financer les aides personnalisées au logement, et l'État en profite, au passage, pour réduire sa contribution. Cet argent va manquer à la construction dans le pays

Je dois en outre rappeler que, si l'article était supprimé, la contribution de l'État au financement des aides personnalisées au logement devrait être rehaussée du même montant. Mais, monsieur le

en lien avec les territoires, et le grand atout d'Action Logement, c'est aussi d'être un acteur au service des territoires. Monsieur le ministre, nous devons travailler ensemble, mais ne préemptons pas le débat. Il serait

est ainsi libellé : La parole est à M. Olivier Cadic. Le 20 mars 2018, dans un discours prononcé à l'Institut de France, Emmanuel Macron se fixait pour objectif de doubler le nombre d'élèves scolarisés dans le réseau d'enseignement français à l'étranger d'ici à 2025.

quels établissements il voudra garantir et à quel taux. Le nouveau dispositif n'a pas été présenté devant l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE), comme cela est prévu pour tout texte intéressant les Français de l'étranger. Le système existant brillamment fait ses preuves depuis 45 ans. L'Anefe instruit les dossiers selon un principe associatif, qui réunit tous les acteurs de l'enseignement français à l'étranger, dont les représentants des parents d'élèves et les élus des Français de l'étranger.

est donc proposé de supprimer l'article 49 et d'étudier, avec les administrateurs de l'Anefe et en prenant l'avis de l'AFE, le système le plus efficient pour progresser dans le sens des ambitions du Président de la République pour l'enseignement français à l'étranger, tout en respectant les règles prudentielles déterminées par Bercy. Quel

possibilité d'octroyer sa garantie aux prêts immobiliers des établissements français d'enseignement à l'étranger. Ce n'est manifestement pas votre objectif,

On ne pouvait pas continuer à octroyer la garantie de l'État, à travers une structure ne répondant pas à la réglementation nationale et européenne, que ce soit, d'ailleurs, pour des questions de monopole bancaire ou pour des questions C'est bien ce système qui met en péril la garantie pour les projets immobiliers des établissements français à l'étranger, et non le nouveau dispositif. Enfin, il est essentiel que le dispositif de garantie réponde aux exigences européennes en matière d'aides d'État ; mais ça, monsieur Cadic, monsieur le ministre, sans respecter les ratios prudentiels et en violation du monopole bancaire. C'est pourquoi nous proposons un dispositif public. L'Anefe continuera à gérer les garanties accordées, à hauteur de 340 ou 350 millions d'euros

Je voudrais dire mon désaccord avec mon collègue Olivier Cadic. Il me semble normal que l'AEFE, qui est la maison mère, en quelque sorte, de tous les établissements d'enseignement français à l'étranger, soit partie prenante à la politique immobilière. Nous avons un plan de doublement du système éducatif français à l'étranger, dans les cinq à dix années qui viennent. L'AEFE sera au coeur de ce dispositif.